La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il était attendu depuis longtemps ! C'était un engagement du Président de la République, et, après bien des difficultés, Franck Riester avait fini par convaincre de le faire inscrire à l'ordre du jour. Pourtant, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, à même d'armer notre audiovisuel, public comme privé, pour lui permettre de relever les défis générés par le nouveau monde, numérique a été abandonné au milieu du gué, en pleine procédure parlementaire. Bien sûr, on peut arguer de la crise sanitaire ; mais, précisément, les conséquences de celle-ci sur les usages et l'accélération observée des mutations en cours dans le secteur audiovisuel n'ont fait que renforcer le besoin de se remettre à jour par rapport à la loi du 30 septembre 1986, texte conçu pour le monde hertzien. Lors du colloque que notre commission avait organisé en juillet 2018, intitulé « Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ? alors que la réforme, celle de la redevance notamment, avait déjà été menée dans leurs pays respectifs, les représentants des audiovisuels publics européens, à comprendre le retard pris chez nous, nous avaient dit attendre beaucoup de la France, jugée comme une référence dans son combat pour l'exception culturelle. Quelle déception !

sur l'avenir de l'audiovisuel et de la création. Je salue à cet égard l'implication forte des sociétés d'auteurs, qui a permis la mobilisation organisée à Bruxelles aux côtés des parlementaires pour faire adopter ces directives. Avec l'abandon de la réforme de la gouvernance, le groupe Union Centriste regrette le retard qui va continuer à être pris alors que la concurrence s'intensifie, que les nouveaux formats et offres se multiplient, que partout le paysage se recompose pour mieux aborder les défis du siècle. L'actualité récente, marquée par le rapprochement de TF1 et de M6, nous le rappelle encore, si besoin était ! Plus encore, nous réprouvons l'abandon de la réforme de la contribution à l'audiovisuel public que Franck Riester avait pourtant promise pour 2021 au plus tard. au plus tard. Cette réforme différée est non seulement nécessaire pour faire évoluer l'assiette d'une redevance devenue injuste, les supports de diffusion ayant considérablement évolué, mais aussi pour prévenir la chute attendue de son rendement. Tout cela, je le disais déjà en 2011 dans un rapport sur l'avenir du financement de France Télévisions, et mes collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin ne disaient pas autrement en 2015. Pour couronner le tout, avec la suppression de la taxe d'habitation, nous n'avons plus aucune visibilité sur une ressource pérenne qui constitue par ailleurs la principale garantie d'indépendance, nécessaire pour développer des projets dans la durée. Franchement, il aurait été raisonnable d'assurer le modèle économique de notre audiovisuel public, qui concerne cinq entreprises et des milliers d'emplois directs et indirects, avant les échéances électorales de l'année prochaine. Vous comprendrez donc que je ne puisse que joindre ma voix à celle de notre rapporteur, dont le constat est alarmant. Bien entendu, nous souscrivons aux dispositions du texte portant création de l'Arcom. loi contient en effet des dispositions fondamentales et attendues afin de mieux lutter contre le piratage et pour la protection des auteurs. Je fais partie des parlementaires qui ont vécu, ici même, les balbutiements d'une législation visant à protéger les auteurs et la création à l'ère du numérique,

il paraît naturel d'améliorer notre législation et de faire évoluer nos autorités de régulation, promises à de plus larges missions. Nous entretenons d'ailleurs des échanges réguliers avec les présidents de ces autorités, ne serait-ce qu'à l'occasion de leur bilan annuel. À plusieurs reprises, les présidents de la Hadopi et du CSA, mais également de l'Arcep et de la CNIL ont été entendus ensemble afin que nous puissions mesurer les convergences et rapprochements souhaitables pour plus d'efficacité. Je profite de cet instant pour saluer le remarquable travail de l'ancien président de la Hadopi, Denis Rapone, dont le mandat parvenait à échéance en janvier dernier. Compte tenu de l'évidence de certaines synergies, je regrette, comme notre rapporteur, que le lien avec l'Arcep ne soit pas sanctuarisé dans ce texte.

sur ce sujet, rappelons que la commission a été précurseur en organisant très tôt des tables rondes sur le piratage sportif et en émettant des propositions fortes. C'est ainsi qu'en commission, avec mes collègues Pierre-Antoine Levi, Michel Laugier et Claude Kern, nous avons souhaité, par nos amendements, compléter utilement le texte initial. S'il y aura, bien sûr, quelques points de divergence entre nos groupes sur certains sujets, je me réjouis que nous nous soyons retrouvés sur un certain nombre de propositions importantes, notamment pour renforcer l'effectivité des droits d'auteur et des droits voisins voisins ; pour faciliter l'accès aux oeuvres et aux catalogues ; pour préserver l'attractivité de la TNT. Sur ce sujet, je vous proposerai d'aller plus loin aujourd'hui en donnant pouvoir à l'Arcom d'autoriser l'utilisation de formats d'images améliorés,

le maintien de France 4. L'ensemble de notre commission s'était mobilisé sitôt l'annonce de sa suppression, entendant défendre la filière du cinéma d'animation, mais surtout une offre publique exempte de toute publicité, s'agissant de la chaîne de l'éducation, de la culture et de la citoyenneté, véritable alternative, pour nos jeunes, aux plateformes commerciales. Alors que, ces dernières années, conseil d'administration après conseil d'administration de France Télévisions, je n'ai cessé de redire l'importance de France 4, je suis heureuse que le Président de la République ait opportunément tranché en faveur de son maintien,

J'en profite pour inviter à la réflexion sur ce qui pourrait être fait en région dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens passés entre les collectivités régionales et les antennes de France 3. Encore une fois, les initiatives prises pendant le confinement méritent d'être pérennisées et développées. Elles permettent notamment de toucher des publics empêchés de se rendre dans les salles de spectacle. C'est cela aussi, la mission de l'audiovisuel public : assurer le respect des droits culturels de chacun.

renforcer les missions des autorités de régulation. Pour ma part, j'étais déjà intervenue en ce sens pour le CSA à la suite du vote de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, mais également à plusieurs reprises en faveur de la CNIL et de l'Anssi, faiblement dotées. Il est vrai que, pour assurer le nécessaire financement de celles-ci, il est fondamental de recouvrer le juste impôt dû par ces plateformes, qui justement favorisent les problèmes que nous devons nous attacher à résoudre, mais qui pratiquent, comme chacun le sait, l'évasion fiscale.

ont permis la disponibilité courante de centaines de chaînes du monde entier. Les nouvelles technologies ont bouleversé les conditions mêmes de la création et de la production audiovisuelles et ont révolutionné les usages, notre paysage de grandes plateformes américaines qui, échappant aux régulations essentielles voulues par les législateurs de 1986, ont contourné les obligations de financement et de fiscalité imposées aux acteurs traditionnels. Elles se sont imposées en chamboulant notre système de financement de la création, la chronologie des médias, mais également les accords existants entre les chaînes de télévision et les producteurs. Cette situation nécessitait au moins que nous en débattions globalement,

révolutionner notre paysage médiatique en le concentrant comme jamais, lui qui l'est déjà tant et trop, face à un audiovisuel public privé de recettes publicitaires

consacrés à l'article 34 de notre Constitution. La première conclusion que nous devons vite en tirer, c'est de renforcer notre audiovisuel public. Face à ce nouveau géant du privé, celui-ci devra avoir les moyens de faire rayonner toutes ses missions d'intérêt général : l'information libre, l'exception culturelle, l'éducation et le financement à un haut niveau de la création. Cela passe par la réforme tant attendue et repoussée de la redevance, qui doit devenir universelle, mais aussi par l'arrêt des baisses budgétaires que ce gouvernement s'est entêté à renouveler année après année, ce malgré les efforts inouïs que les sociétés de l'audiovisuel public et leurs personnels ont consentis depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je ne peux que me réjouir que le Président de la République ait enfin renoncé à supprimer France 4,

que chacun le sait, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de convaincre de la nécessité du maintien de cette chaîne de la jeunesse en proposant d'y revenir à chaque débat, comme lors du dernier budget. seul au début avec mes collègues socialistes, puis nous avons été utilement rejoints par la commission dans son ensemble. Jusqu'à hier, on nous opposait une logique comptable. C'est une victoire, qui doit nous encourager à ne jamais rien lâcher quand la cause est juste, même lorsqu'on nous dit qu'il n'y a plus rien à faire.

loi aussi fondatrice que celle de 1986 pour moderniser la réglementation à l'heure du numérique, sans pour autant remettre en cause les principes de cette loi de 1986, à savoir la nécessaire régulation et l'aide à la création, essentielle pour maintenir notre exception culturelle.

À l'heure de la révolution numérique, cantonner le CSA au contrôle et à la régulation de la télévision ainsi que de la radio, en laissant la diffusion audiovisuelle sur internet sans réelle instance de contrôle et de régulation, était un contresens.

par la droite sénatoriale, qui a intégré une transaction pénale en remplacement du dispositif actuel de réponse graduée. En tout état de cause, le piratage du sport est symptomatique du problème.

C'est pourquoi je me suis permis d'en profiter pour poser plus globalement la question de la diffusion du sport à la télévision en vous proposant plusieurs des préconisations du rapport que j'ai remis au Gouvernement il y a quatre ans, car il semblait faire consensus. Excellent rapport ! Elles concernent la diffusion gratuite d'événements majeurs, la diffusion du sport féminin et du handisport. Le Gouvernement a aussi décidé d'aborder dans ce texte de loi le sujet des reventes de catalogues. Cette mesure est nécessaire, et nous la soutiendrons en lui sa force initiale. Il est important de protéger les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises. Le risque existe surtout pour les ventes à des acteurs étrangers qui n'ont pas la même exigence que nous quant à notre patrimoine. Nous regrettons que la stratégie choisie finalement, à la suite de la décision du Conseil d'État, soit si molle. Nous tenons à une version plus contraignante. C'est pourquoi nous avons amendé le texte en ce sens. Enfin, à l'heure où les négociations entre Google et les éditeurs et agences de presse sur l'application de la loi que j'ai initiée concernant les droits voisins de la presse, et dans l'attente également d'une décision de l'Autorité de la concurrence, j'ai souhaité, avec le soutien unanime de la commission, dont je remercie tous les acteurs,

J'espère que ces améliorations bénéfiques pour le secteur que nous défendons seront adoptées et maintenues jusqu'au vote définitif du texte et qu'elles ne seront pas détricotées par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. La parole est

c'est la déception qui prédomine. Comment un texte annoncé, attendu, peut-il passer sous silence l'essentiel, c'est-à-dire les enjeux liés aux affrontements concurrentiels dans le paysage audiovisuel ? Le Gouvernement justifie son inaction par la crise sanitaire. Pourtant, l'engouement suscité durant cette période par les plateformes américaines a bien montré l'urgence de défendre l'ensemble de la chaîne de création audiovisuelle française.

Je m'alarme plus particulièrement pour l'audiovisuel public, dont il faudra bien un jour moderniser l'offre, revoir les moyens et repenser l'organisation ainsi que la gouvernance. Nous prônons depuis plusieurs années, au Sénat, la création d'une société mère unique, à même de définir une stratégie globale et d'affirmer une identité spécifique. L'audiovisuel public doit plus que jamais se concentrer sur ses missions et marquer sa différence. C'est ce modèle d'une « BBC à la française » qu'envisageait le rapport de nos collègues Leleux et Gattolin en 2015. Le premier projet de loi, malheureusement avorté, en reprenait les conclusions essentielles. Il n'en est, hélas ! aujourd'hui plus question. Il est donc bien clair que le Gouvernement a renoncé à traduire dans la loi l'engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron pour l'audiovisuel public. Il ne souhaite pas davantage s'impliquer sur des projets susceptibles de faire débat dans le paysage audiovisuel privé. Bref, le projet de loi gouvernemental est maigrelet : création de l'Arcom, adaptation de la lutte contre le piratage, contrôle de la cession de catalogues d'oeuvres françaises. Certes, ce sont là quelques mesures utiles, mais bien limitées dans leur ampleur. Fort heureusement, désormais dans ce texte des propositions ambitieuses de notre rapporteur Jean-Raymond Hugonet, qui y a introduit plusieurs marqueurs essentiels. Concernant l'audiovisuel public, notre rapporteur a proposé qu'une des chaînes du groupe France Télévisions soit consacrée à des programmes dédiés à la jeunesse. Le Sénat est ainsi fidèle à sa volonté de pérenniser France 4, que le Gouvernement voulait fermer en août. Nous pouvons nous féliciter, cher Jean-Raymond Hugonet, que le Président de la République se soit finalement rallié à notre position il y a trois jours, en retenant précisément notre formule de programmation jeunesse en journée et culturelle en soirée.

Plusieurs années de pratique de « réponse graduée » nous montrent combien il est nécessaire de responsabiliser davantage les internautes. Notre commission a également veillé à la protection des droits d'auteur dans le contexte d'utilisation des contenus par les plateformes. Je pense, notamment, aux accords que nous souhaitons voir conclure avec le secteur de la presse. Nous écouterons attentivement vos remarques sur ce sujet, madame la ministre. Enfin, notre rapporteur propose de rééquilibrer les rapports entre distributeurs et producteurs. C'est nécessaire, car les chaînes françaises sont aujourd'hui contraintes de financer des programmes dont elles ne maîtrisent pas les droits par la suite, et elles ne peuvent ni contrôler leur revente à des concurrents ni en attendre de recettes. Or le contrôle de l'exploitation des oeuvres dans un environnement désormais mondial devient déterminant pour les ressources des chaînes et, donc, pour leur capacité à rester des opérateurs forts du financement de la création. Nous espérons que les propositions de notre rapporteur seront finalement entendues et marqueront l'architecture définitive du texte, sachant, par ailleurs, que nous avons toute confiance dans la négociation professionnelle entre les acteurs. À la suite des travaux de notre commission et des propositions de notre rapporteur, ce projet de loi, largement amendé, a donc pris une nouvelle dimension. Aussi le groupe Les Républicains lui apportera-t-il tout son soutien. La parole est

ces derniers mois, plusieurs big-bangs annoncés par le Gouvernement se sont transformés en mesurettes. Concernant l'audiovisuel, ce sont les aléas épidémiques et calendaires qui ont eu raison du projet de loi structurel que notre assemblée aurait dû examiner. À défaut, c'est un texte à l'épure plus limitée qui nous est présenté. Pourtant, la covid n'a pas eu raison du piratage et n'a pas fait disparaître les attentes d'un secteur audiovisuel constitutif de notre patrimoine commun. À rebours de ce qui se fait habituellement à cette tribune, je tiens à souligner ce que ce projet de loi ne dit pas, ne crée pas et ne prévoit pas, en dépit des bouleversements induits par la société de l'écran. Les enjeux du numérique impliquent, en effet, de faire évoluer un cadre législatif et normatif par trop dépassé. Nous pensons aux lois de 1986 et 2009, mais également aux instruments qui assurent actuellement la régularisation qu'une grande nation culturelle doit à ses créateurs. Cette déception sur le cadre restreint de la loi se double d'une inquiétude légitime, car les crédits de l'Arcom dépendront d'un budget dont nous ne savons rien et qui, cette année, revêtira deux caractéristiques particulières. Il s'agira de la dernière loi de finances de ce quinquennat et celle-ci s'inscrira dans un contexte de crise dont nous savons la rudesse pour le monde culturel. J'insisterai sur trois éléments du projet de loi originel que notre rapporteur et plusieurs de mes collègues ont eu à coeur de gommer. Le texte initial ne traitait pas, hélas ! des disparités réglementaires qui obèrent les capacités d'investissement des acteurs historiques. Je pense au dispositif anti-concentration mentionné à l'article 41 de la loi Léotard, dont le CSA estime lui-même qu'il est obsolète face aux évolutions démographiques, économiques et technologiques du secteur. Je pense aussi aux limites imposées aux groupes en matière de rachat des chaînes de la TNT et au manque d'incitations à l'intégration verticale indispensable au financement de programmes de flux, qui contribuent également au dynamisme de la création française. Le texte initial ne traitait pas non plus, hélas ! des difficultés d'un secteur radiophonique en crise structurelle, alors que nous célébrons les cent ans de ce média et les quarante ans de la libération de la bande FM. Nous aurions pu intégrer à nos discussions la question du régime des mentions légales ou des quotas. En effet, le développement des plateformes de audio, qui échappent à cette régulation, devra nous conduire tôt ou tard à répondre à un dilemme fondamental : étendre ces quotas au service de musique à la demande ou réviser les trois régimes existants. Nous savons que l'enchevêtrement des critères bride parfois la liberté éditoriale des professionnels. Le texte initial ne traitait pas non plus, hélas ! de la modernisation d'une TNT que nous savons économique, écologique et surtout vectrice d'un maillage territorial indispensable à l'égalité devant l'offre audiovisuelle. En somme, nous débattons principalement d'une loi antipiratage, dont la mesure phare demeure la création de l'Arcom. Sur ce point aussi, pourquoi ne pas être allée plus loin, madame la ministre, en vous inspirant du modèle britannique et de son puissant office des communications ? Je rappelle que, chez nos voisins, qui ont eu plus de dix ans d'avance sur la directive SMA, ce sont cinq entités fusionnées et des capacités d'enquête qui garantissent l'effectivité des missions de cette super-autorité de contrôle. Madame la ministre, c'est avec la saine exigence qui caractérise cette assemblée, son esprit d'ouverture et sa technicité que nous saluons les intuitions d'un texte dont le cadre nous apparaît toutefois trop restreint. Permettez-moi de citer l'un de vos illustres prédécesseurs pour vous dire notre bienveillante déception et l'esprit constructif qui nous guide, sous l'impulsion du rapporteur Hugonet. Ainsi que l'écrivait Maurice Druon, « la critique nous est profitable, quand elle nous aide à travailler dans le sens de l'amélioration

je tiens tout d'abord à saluer la capacité d'écoute, la capacité de dialogue et la qualité des travaux de notre rapporteur. J'ai souhaité, madame la ministre, chers collègues, cibler mon intervention sur l'article 3 de ce projet de loi, qui traite de la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct. Le piratage des compétitions sportives est un véritable fléau et une réelle menace pour l'écosystème sportif français. Les pertes s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros pour les diffuseurs et les ayants droit, et le phénomène est en pleine croissance. Cette menace est également directe pour le sport amateur, qui bénéficie- je le rappelle -des retombées de la taxe Buffet, mécanisme de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Les récents déboires relatifs aux droits TV du football ont un peu plus fragilisé l'écosystème. C'est pourquoi il est important de renforcer le soutien à ce secteur. Aujourd'hui, il est plus que jamais indispensable d'adapter le cadre juridique existant aux spécificités et aux nouveaux défis que pose le piratage sportif. Je tiens à rappeler ici l'engagement de longue date, comme l'a souligné notre collègue Catherine Morin-Desailly, du Sénat sur ce sujet. Une première étape a été franchie à l'occasion de l'adoption de la loi du 1 mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. L'article 24 de cette loi, adopté ici au Sénat, encourage les acteurs du sport et du numérique à négocier la conclusion d'accords de bonnes pratiques de lutte contre le piratage. C'est dans ce cadre que s'est créée l'Association pour la protection des programmes sportifs, qui regroupe ayants droit et diffuseurs. Toutefois, ce dispositif s'avère à ce jour insuffisant. Après plusieurs mois de dialogue entre professionnels, il est désormais nécessaire que des mesures législatives viennent renforcer les dispositifs protégeant les ayants droit et diffuseurs et assurent une lutte enfin effective contre le piratage de contenus sportifs en direct. Le dispositif proposé par le Gouvernement au travers de ce texte a pu faire naître quelques inquiétudes, notamment à l'alinéa 12. Il est regrettable qu'après l'examen de deux dispositifs un troisième mécanisme ait été présenté, avec une rédaction différente. Lors de l'examen en commission, plusieurs amendements sont venus renforcer le dispositif initial, notamment en centralisant le contentieux du piratage des retransmissions sportives en direct auprès du tribunal judiciaire de Paris. En prévoyant que la durée de l'ordonnance dynamique portera sur douze mois au maximum,

la rédaction de l'alinéa 12 de cet article 3. J'espère que ces avancées, largement travaillées avec les ayants droit et les diffuseurs, qui sont les victimes de ce piratage, seront retenues par la majorité à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, je souhaite que ce texte soit rapidement adopté pour entrer en action au plus vite. Après plus d'un an de crise sanitaire, ce soutien apporté aux acteurs est largement attendu. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que nous avons adopté en commission un article permettant à la Hadopi de mettre en oeuvre dès la promulgation de cette loi les dispositifs relatifs à la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, sans attendre la création de l'Arcom, qui devrait intervenir trois mois après la promulgation du texte. Là encore, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien, madame la ministre, afin de permettre à ce dispositif d'être effectif dès la saison sportive prochaine, à la rentrée de 2021.

amendement vise à élargir la portée de la mission pédagogique attribuée à l'Arcom en matière de protection des oeuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou des droits d'exploitation audiovisuelle. Le projet de loi tel qu'il est présenté ne cible aujourd'hui que les publics scolaires. Pour que cet objectif soit adressé au bon public et que la nouvelle autorité remplisse avec efficacité son objectif de sensibilisation à la diffusion de l'offre légale, il apparaît utile d'étendre expressément cette mission aux élèves de l'enseignement supérieur, eu égard à leur intense usage tant professionnel que personnel des contenus à protéger. La création de l'Arcom, qui pérennise une réponse graduée saluée pour son caractère pédagogique, offre l'occasion de gagner en efficacité quant au ciblage des publics directement concernés par le piratage. de la commission ? Cet amendement part du constat, tout à fait juste, d'un manque de connaissances par les étudiants des grands axes de la propriété intellectuelle. C'est d'autant plus vrai que les étudiants actuels sont issus d'une génération confrontée

Je suis bien sûr favorable sur le fond à l'extension des actions de sensibilisation en direction des étudiants, mais le texte le permet déjà expressément puisque

de pouvoir informer les internautes adultes sur les risques encourus en cas de téléchargement illicite et les sensibiliser à l'existence d'une offre légale. Je suis défavorable à cet amendement, non sur le fond, mais en raison des effets contreproductifs qu'il pourrait avoir. Je ne veux pas faire de peine à l'auteur de l'amendement, mais je peste déjà suffisamment contre les injonctions de notre assemblée

de plateformes, plus les contenus seront éclatés et plus les coûts seront élevés : 10 euros pour OCS, 8 euros pour Netflix, 6 euros pour Amazon Prime, 7 euros pour Disney+ et Salto, sans parler des 22 euros nécessaires pour accéder au contenu de Canal+. La facture monte très vite pour accéder à ces films et séries. En ce qui concerne la musique, même si YouTube dispose d'une bibliothèque importante pour les chaînes officielles d'artistes, le constat est malheureusement le même. Il me semble donc qu'il y a un travail à mener en ce sens, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que, comme je l'ai sous-entendu à l'instant, c'est le meilleur outil contre le piratage et, deuxièmement, parce que le fonctionnement actuel et la difficulté croissante d'accéder au contenu culturel à éloigner les personnes les plus fragiles économiquement de la culture. Or, comme le rappelait l'Unesco au début de cette crise sanitaire, la culture est un bien commun essentiel et source de résilience. Au moment où la santé psychique des Françaises et des Français est durement éprouvée par la crise et la diminution des interactions sociales, la culture prend une une importance encore plus grande. C'est pourquoi il nous semble nécessaire de confier à l'Arcom une mission sur l'accessibilité, notamment financière, et le développement de l'offre légale. Quel est l'avis de la commission ? Les auteurs Les auteurs de cet amendement veulent attirer l'attention sur un aspect essentiel des offres numériques pour les oeuvres audiovisuelles, qui est leur caractère fragmenté. En effet, si l'on veut aujourd'hui bénéficier de l'ensemble des oeuvres, il faut multiplier les abonnements, ce qui s'avère excessivement onéreux. Par comparaison, l'offre de musical légale est parvenue, sur quelques plateformes, à concentrer toute l'offre, ce qui n'est pas étonnant de la part des musiciens. musiciens. Il n'est pas certain que l'Arcom ait réellement les moyens ou la vocation de lutter contre ce qui est une conséquence de l'explosion des coûts de production dans une industrie largement mondialisée, ni que son rôle en la matière puisse être utile. La commission a donc émis un avis défavorable. Quel est Même avis, pour les excellentes raisons exposées par M. le rapporteur.

par les producteurs leur engagement en matière de blocage technique. Vous achetez un DVD et vous souhaitez en faire une copie numérique pour votre usage personnel ? Dans la majorité des cas, vous ne pourrez pas extraire le DVD malgré votre droit à la copie privée du fait du blocage technique. Vous pensez acheter un jeu vidéo sur une plateforme de type Steam ? Vous n'achetez en fait que le droit d'y jouer. Les utilisateurs des plateformes Sony peuvent témoigner du stress de voir une vidéothèque disparaître après l'annonce des fermetures des boutiques PS3 et PS Vita. Enfin, si vous achetez de la musique sur une plateforme de type iTunes, je vous souhaite bien du courage pour trouver le fichier dans votre ordinateur ... Cet amendement vise donc à confier à l'Arcom une mission de protection des droits des acheteurs de contenus. La lutte contre le piratage ne pourra passer que par une relation de confiance entre les acteurs culturels et les consommateurs, mais cela implique que ces derniers puissent jouir pleinement de leurs droits, une fois qu'ils ont acheté un contenu. Quel est l'avis de la

Je formulerai les mêmes remarques de fond que celles que j'ai émises sur les précédents amendements. Le code de la propriété intellectuelle confie d'ores et déjà à la Hadopi une mission de régulation des mesures techniques de protection

que leur contribution à la création artistique et culturelle ». En l'état, la France a pris un retard dommageable, même si tous les secteurs ne sont pas concernés de la même manière. Pour ne prendre que l'exemple de la télévision, la proportion de programmes qui doit comprendre un sous-titrage dépend directement de l'audience de chaque chaîne. Les chaînes dont la part d'audience est inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision doivent sous-titrer l'ensemble de leurs programmes, tandis que pour les chaînes hertziennes dont l'audience est inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision une convention conclue avec le CSA fixe les proportions des programmes accessibles. S'il ne faut pas omettre les difficultés techniques réelles pour les éditeurs, nous devons passer un nouveau cap en matière d'accessibilité et d'inclusivité. Comme l'a montré cette crise sanitaire, les oeuvres culturelles sont essentielles. On en était déjà persuadé, mais nous avons eu devant les yeux les conséquences néfastes d'une disparition de la culture dans notre quotidien. D'ailleurs, si le dernier rapport du CSA sur la représentation du handicap à l'antenne et l'accessibilité des programmes de télévision aux personnes handicapées montre des progrès, ces derniers sont largement insuffisants et surtout inégalement répartis selon les éditeurs. Il est donc essentiel de renforcer cette mission. Quel qu'aux éditeurs, qui devraient rendre l'ensemble des contenus accessibles, c'est-à-dire leur appliquer le sous-titrage, l'audiodescription et l'adaptation chromatique. On ne peut que saluer cette tant elle traduit la volonté de donner toute leur place aux publics handicapés. Je rappelle d'ailleurs que le 26° du paragraphe I de l'article 1 confie déjà au régulateur la responsabilité de veiller au respect par les éditeurs de livres de l'exception « handicap », en lien avec la Bibliothèque nationale de France. me semble que cette idée, appliquée à l'audiovisuel, pourrait se heurter à des considérations de coût, si l'ensemble des oeuvres devait bénéficier des mesures d'accessibilité. Il n'est pas certain qu'une approche aussi radicale soit économiquement viable. En tout cas, elle

Je ne peux que constater avec vous que l'accessibilité aux programmes pour les publics handicapés mérite de progresser- les excellents rapports du CSA le montrent abondamment.

d'assurer la garantie effective de l'exception au droit d'auteur prévue par la loi au profit des personnes en situation de handicap, et le projet de loi prévoit de renforcer les pouvoirs de l'Arcom sur ce sujet à travers la possibilité qui lui sera reconnue de mettre en demeure les éditeurs de respecter leurs obligations légales. L'un de vos arguments est donc d'ores et déjà satisfait. Par ailleurs, la loi confie au CSA le soin de veiller à l'accessibilité des programmes télévisés aux personnes handicapées par le sous-titrage, la langue française des signes ou l'audiodescription. Le CSA s'assure annuellement que les chaînes remplissent leurs obligations en matière d'accessibilité des programmes et rend compte de ce contrôle dans un rapport public. En réunissant les pouvoirs de la Hadopi et du CSA sur ce sujet, l'Arcom sera en mesure d'agir en faveur d'une plus grande accessibilité des oeuvres. Ainsi, l'objectif que vous portez est d'ores et déjà satisfait, car il est de fait

L'amende transactionnelle risque de surcroît de pénaliser les internautes les moins renseignés : ceux-ci paieront par crainte d'un procès, alors que ceux qui sont le plus au fait des choses estimeront plus facilement que le risque d'être condamné est faible. Enfin, elle ne permet aucune distinction en fonction du volume de téléchargement ou d'éléments qui pourraient être considérés comme des circonstances atténuantes par la justice.

Dans la vie réelle, la loi dite Hadopi ne s'attaquera, de fait, qu'aux plus novices, ceux qui ne savent pas masquer leur adresse IP. Les véritables délinquants seront épargnés, car ils connaissent les moyens technologiques d'échapper à la surveillance. » Dix ans plus tard, avec l'émergence des VPN, c'est encore plus vrai.

On renforce la lutte contre le piratage et les moyens des services audiovisuels contre les nouveaux entrants sur le marché, mais rien n'est fait pour améliorer concrètement l'accès aux contenus culturels, ce qui, pourtant, a longtemps fait la fierté et la spécificité de la France dans le cadre de l'exception culturelle, vue comme un outil au service de la Nation. La parole

qui captent des revenus considérables avec leurs pratiques illégales au détriment des créateurs et titulaires de droits sportifs. Nous ne souhaitons pas, en revanche, modifier l'équilibre de la réponse graduée, qui se veut un outil au service de la prévention et de la pédagogie. Lorsque la pédagogie ne suffit pas, la réponse graduée peut conduire à des sanctions judiciaires, sous l'autorité d'un juge, mais nous ne voulons pas aller plus loin dans la sanction des internautes,

des auteurs de faits délictueux. J'entends les arguments qui ont été avancés : il ne faut pas pénaliser les internautes les moins renseignés ; cette amende s'apparente à un droit de pirater ; la philosophie de la loi est de sanctionner plutôt les sites pirates, etc. Je veux simplement dire que nous parlons ici non pas d'une piraterie occasionnelle, mais d'internautes déjà prévenus trois fois, donc relativement avancés dans leur comportement délictueux. Il est absolument anormal, quel que soit le domaine, qu'une violation de la loi ne soit jamais sanctionnée ! Il me semble que la transaction pénale, un mécanisme équilibré très attendu par les ayants droit, s'inscrit très logiquement comme la dernière étape d'une réponse pédagogique. Elle est tout à fait complémentaire des actions prévues dans le présent article pour sanctionner les sites eux-mêmes, qui ne vivent d'ailleurs qu'en raison de l'appétit de certains pour le piratage.

les administrations, les entreprises pourraient être incitées à limiter au maximum la mise à disposition d'un accès internet au profit de leurs agents ou de leurs usagers

à elle la formulation « service [ ...] dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu » du service original. Le présent projet de loi revient à la rédaction de la loi Avia.

et identique du site originel. C'est ce que l'on peut retrouver dans les sites strictement identiques qui réapparaissent grâce à un simple changement d'extension. En l'espèce, le projet de loi va bien plus loin et, surtout, laisse à l'autorité administrative le soin de placer le curseur. Est-ce qu'un site qui changerait la colorimétrie d'un film piraté, son rythme ou son montage serait considéré comme le site miroir de n'importe quel site de piratage bloqué par décision judiciaire ?

Le projet de loi prévoit que l'Arcom pourra demander aux intermédiaires techniques d'empêcher l'accès aux sites miroirs. Il ne fait pas de doute que cette rédaction vise notamment les fournisseurs d'accès à internet. En revanche, il n'est pas certain que les moteurs de recherche soient visés, dès lors que ceux-ci ont pour mission non pas de donner accès à des sites, mais seulement de les référencer. Or il me paraît absolument indispensable que l'Arcom puisse également s'adresser à ces acteurs. L'amendement du Gouvernement vise donc à ne laisser aucun doute quant à la possibilité pour cette autorité de demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites miroirs.

d'ailleurs enrichi en commission par les amendements de nos collègues Michel Laugier et Pierre-Antoine Levi, me paraît au contraire fondamental, compte tenu de l'évolution des formes de piratage. En ce qui concerne la caractérisation de ces sites, jugée par les auteurs de l'amendement imprécise, j'avoue avoir eu la même préoccupation au début de mes travaux, aux avantages d'une formulation suffisamment large : elle permet notamment de prévenir tout risque de contournement. Je rappelle d'ailleurs que les sites qui s'estimeraient injustement fermés auront toute latitude pour contester cette décision devant les tribunaux. La commission est donc défavorable

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d'injonction dynamique permettant aux titulaires de droits sur les oeuvres protégées et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une décision judiciaire de saisir directement toute personne susceptible de contribuer à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin,

Force est en effet de constater que le dispositif prévu par le projet de loi, qui nécessite le passage par l'autorité administrative et dont il n'est pas avéré qu'il sera le plus souvent suivi d'effet compte tenu de la possible localisation du contrefacteur en dehors de l'Union européenne, ne peut constituer le seul moyen d'assurer l'efficacité des mesures judiciaires prononcées. Il importe que les bénéficiaires d'une décision judiciaire ordonnant des mesures ayant pour objet de faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin soient également en situation de répliquer dans un temps numérique aussi rapide que celui des contrefacteurs.

En revanche, s'agissant des cas plus complexes de lutte contre les sites miroirs, son expertise technique et sa légitimité pourraient contribuer au traitement des difficultés rencontrées. La mesure proposée par le présent amendement est attendue par l'ensemble du secteur culturel, que ce soit le cinéma, l'audiovisuel, le livre ou la musique. C'est la raison pour laquelle, malgré un avis défavorable du rapporteur en commission, j'ai souhaité déposer cet amendement en séance pour que Mme la ministre puisse s'exprimer sur ce sujet. L'amendement Nous avons déjà débattu en commission de l'intérêt de mettre en place un mécanisme supplémentaire de lutte contre le piratage, dit « injonction dynamique ». Un tel dispositif aurait l'immense avantage, en théorie, de rendre la procédure de blocage des sites plus rapide, plus rapide, en établissant un lien direct entre l'ayant droit et le fournisseur d'accès. Il concernerait les mêmes services autrement accessibles ou localisés, selon ses propres Le juge autoriserait, dans la décision initiale, l'actualisation de sa mesure. Si un site identique apparaissait, les ayants droit saisiraient directement le prestataire, qui aurait l'obligation de bloquer le site ; sa responsabilité serait alors dégagée. Comme je le soulignais en commission, l'injonction dynamique serait en réalité une procédure concurrente de celle mise en place par le présent article pour lutter contre les sites miroirs, avec cependant deux différences. D'une part, la procédure « sites miroirs » est plus large, puisqu'elle ne concerne pas uniquement les sites identiques, mais également les sites qui reprennent les contenus de manière substantielle. Dans le cas de l'injonction dynamique, le site doit être rigoureusement identique, seule l'adresse étant changée. D'autre part, l'injonction dynamique fait l'économie du passage par le filtre de l'Arcom, en mettant en relation directe les ayants droit et les fournisseurs d'accès. Cela présenterait le mérite de la rapidité, selon les auteurs de cet amendement. de cet amendement. J'y vois surtout l'inconvénient de priver le futur régulateur d'une extension de ses compétences, alors que l'objet même du projet de loi est de le renforcer et de le conforter. Compte tenu du nombre de personnes potentiellement concernées parmi les ayants droit, le filtre de l'Arcom est utile pour éviter que les prestataires soient submergés de demandes faites sans concertation. D'ailleurs, j'observe que, même dans le cadre du piratage sportif, il revient à l'Arcom, selon l'article 3 du projet de loi, de jouer le rôle de filtre. Pour résumer, je crois qu'il serait regrettable de vider, dès l'origine, une nouvelle et importante compétence de l'Arcom d'une partie de sa cohérence, sous le prétexte, qui n'est pas avéré, d'un manque de rapidité. Les procédures de blocage seront d'autant mieux appliquées et exécutées qu'elles paraîtront légitimes et fondées. L'Arcom me paraît être le bon outil à cet égard. Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable sur cet amendement. Madame la sénatrice, je partage tout à fait l'argumentation qui vient d'être développée par votre rapporteur. La différence d'approche entre votre proposition et celle du projet de loi tient à votre souhait de faire l'économie du passage par le filtre de l'Arcom, en mettant en relation directe les ayants droit et les intermédiaires techniques pour une meilleure efficacité. C'est ce que vous appelez l'injonction dynamique. Le Gouvernement est extrêmement attaché à la garantie que représente l'intervention de l'Arcom dans la lutte contre les sites miroirs : elle permet, d'une part, d'apprécier le fait qu'un site signalé constitue bien le miroir d'un site bloqué, d'autre part, de notifier la demande de blocage de ce site miroir aux intermédiaires concernés, notamment les fournisseurs d'accès. C'est un point d'équilibre important et il me semble

apparu sur les plateformes de musical voilà quelques années, et se présente sous la forme d'une demande de rapport pour contourner le couperet de l'article 40. Ces fausses connexions sont réalisées soit par des robots ou des logiciels, soit par des « fermes à clics employant à l'étranger des personnes physiques. Elles se font soit à partir d'un nombre démultiplié de faux comptes temporaires, soit le de comptes existants peu utilisés par leur titulaire. En augmentant artificiellement les écoutes et les vues sur les plateformes de, la manipulation de a pour effet de capter indûment des rémunérations revenant à d'autres ayants droit et de fausser la visibilité des oeuvres comme l'appréciation du public. Ces comportements frauduleux relèvent donc de l'infraction d'escroquerie et sont susceptibles de porter préjudice à l'ensemble de la chaîne de valeur : créateurs, producteurs, plateformes et utilisateurs. Si rien n'est fait, ils risquent d'affaiblir à terme le modèle du, qui porte en lui la renaissance économique du secteur. La particularité de la manipulation de est sa capacité d'adaptation permanente aux pare-feux des plateformes et à la veille des ayants droit par le biais de leur distributeur. L'action de ces derniers est par ailleurs limitée, puisqu'ils n'ont de vision que sur leur propre catalogue. C'est pourquoi le rapport envisagé dans le présent amendement pourrait avoir pour triple objectif de dresser le constat de ces pratiques, d'évaluer la possibilité de confier à l'Arcom un rôle de tiers de confiance et d'enquêteur recueillant toutes les données utiles, notamment de la part des plateformes de musical audio et vidéo, d'évaluer les conditions dans lesquelles les plateformes pourront tirer toutes les conséquences du constat préalablement dressé par l'Arcom en vue de remédier aux comportements frauduleux. de la commission ? Cet amendement concerne les faux, c'est-à-dire la capacité de certains à influencer le nombre d'écoutes qui sert de base à la rémunération des artistes. Comme vous le savez, la musique est chère à mon coeur. Aussi, ce sujet me préoccupe, car il remet en cause l'équité entre acteurs. Il existe plusieurs solutions à ce problème. L'une d'entre elles serait de mettre en place ce que l'on peut appeler un modèle centré sur l'utilisateur- en bon français -, où chacun ne rémunérerait que les artistes qu'il écoute réellement, par opposition à la répartition au nombre d'écoutes. Je sais que les principales plateformes étudient actuellement cette question et je milite pour une solution rapide. En ce qui concerne l'amendement, je suis à ce stade sceptique sur la capacité de l'Arcom à jouer un rôle en la matière

par l'orientation du rapport que vous demandez au Gouvernement d'élaborer. Vous souhaitez qu'il étudie l'opportunité de confier à l'Arcom une mission de contrôle et de tiers de confiance en matière de lutte contre les manipulations d'audience.

ailleurs, la question des manipulations d'audience renvoie à un enjeu de répartition des revenus qui ne relève pas non plus des missions de l'Arcom- financement de la création, lutte contre le piratage, promotion de la diversité culturelle ...

national de la musique (CNM). Cet établissement public doté par la loi d'une mission d'observation de l'économie de la filière musicale me semble être l'instance adaptée pour discuter de ces questions qui intéressent tous les acteurs de la musique.

loi LCAP, sur la juste rémunération des artistes auteurs d'arts visuels, graphiques et photographiques pour l'exploitation de leur oeuvre par les plateformes numériques. Pour la première fois en 2016, le Sénat avait posé le principe d'une rémunération équitable. Malheureusement, du fait de sa complexité, le système s'est révélé inopérant et, donc, inefficace pour permettre aux artistes auteurs de bénéficier du fruit de leur oeuvre. C'est pourquoi, en commission, j'ai proposé un nouveau dispositif qui s'inspire des recommandations du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, émises dans le cadre de sa mission sur les services automatisés de référencement d'images. Plus précisément, il prévoit un régime de gestion collective des droits d'auteur étendu, conforme aux exigences européennes et adapté à la situation des auteurs concernés.

car la question de la rémunération des artistes auteurs d'arts visuels, graphiques et photographiques dérivant de l'exploitation de leur oeuvre par les services de référencement constitue un enjeu non seulement concret, mais aussi éthique et politique. C'est un enjeu concret dans la mesure où la situation économique et sociale de ces artistes est périlleuse. Leur précarisation et leur paupérisation,

ailleurs, il ne s'agit ni plus ni moins que d'obliger les plateformes numériques à respecter pleinement le droit d'auteur. L'article 2 A s'inscrit dans le prolongement de ce combat éthique et politique plus global qui vise à faire entrer l'économie numérique dans le droit commun.

À la suite de Mme la sénatrice Sylvie Robert, je souhaite m'exprimer sur ce sujet particulièrement important. Les moteurs de recherche d'images présentent aux utilisateurs un nombre considérable d'images indexées par leurs soins sur les réseaux numériques. Le partage de la valeur liée à l'utilisation en ligne de ces images couvertes par le droit d'auteur suscite des débats depuis plusieurs années. Les tentatives de négociation avec les services de référencement n'ont pas abouti, à ce jour, à un accord qui garantirait une juste rémunération des auteurs.

pouvait être assurée par l'intermédiaire d'une licence collective étendue, ce que prévoit désormais l'article 12 de la directive sur le droit d'auteur. Tel est le sens de l'article 2 A, qui a été introduit dans le projet de loi par la commission de la culture. Au-delà du mécanisme juridique créé par cet article, c'est le message politique envoyé qui est primordial. Ce message est aussi celui du Gouvernement : des solutions contractuelles garantissant une juste rémunération de l'ensemble des créateurs concernés doivent être trouvées, et ce rapidement.

Le Gouvernement qui fait sien cet engagement en faveur de la juste rémunération des créateurs continuera de suivre attentivement l'évolution de la situation au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

du droit exclusif des entreprises de communication audiovisuelle selon la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006. Ce mécanisme de licence légale appliqué aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle garantira une rémunération effective des radios et des télévisions en cas de diffusion de leurs contenus dans les lieux publics accessibles sans paiement d'un droit d'entrée. Aujourd'hui, ces éditeurs en sont privés, contrairement aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes.

mais nous pourrions aller plus loin : la révolution numérique à laquelle nous assistons a fait émerger des pratiques qui s'appuient sur les failles de notre droit de la propriété intellectuelle pour se capter de la valeur, en l'occurrence les contenus des éditeurs, sans que ces derniers en soient informés. Cet amendement tend à ce que l'autorisation accordée au titre du droit de reproduction soit requise au préalable et pour tous types de supports.

Je pense notamment aux programmes des radios qui sont conservés sous la forme de podcasts et rendus disponibles, non seulement sur le site ou l'application du média, mais également sur d'autres, comme. Cet article précise que l'autorisation de l'éditeur est requise pour l'utilisation de ces programmes, en direct comme en différé. Cette disposition constitue un progrès incontestable.

Plus important, leur adoption aurait pour effet de conditionner au paiement d'une redevance la diffusion du programme d'une radio ou d'une télévision dans un lieu ouvert au public, comme un salon de coiffure ou un événement retransmis par une collectivité.

n° 7 rectifié. En raison de l'évolution technologique, les entreprises de communication audiovisuelle, comme les éditeurs de services de radio et de télévision, effectuent aujourd'hui, de manière quasi systématique, la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes propres avant diffusion et sont, à ce titre, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au sens des articles L. 213-1 et L. 215-1 du code la même évolution des technologies et des supports d'enregistrement, on constate une hausse des copies de contenus. De plus en plus, en effet, les utilisateurs consomment, téléchargent et enregistrent les programmes sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Afin de compenser la perte subie par les titulaires de droits voisins que sont les éditeurs de radio et de télévision par suite de ces reproductions, le présent amendement vise à confirmer expressément qu'ils bénéficient du dispositif de rémunération pour copie privée, au même titre que les actuels bénéficiaires du système. Cette modification est conforme à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui permet, voire impose, cette extension de rémunération pour copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle.

Monsieur le sénateur, je tiens à saisir l'occasion qui m'est donnée pour saluer votre engagement depuis plusieurs années en faveur de la consécration d'un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse et, plus largement, en faveur de la défense des créateurs. Il fallait que cela soit dit.

Les plateformes numériques qui captent la valeur créée par les journalistes, les éditeurs et les agences doivent contribuer au financement de ce secteur. Nous savons tous que la mise en oeuvre de ce droit se heurte malheureusement à des difficultés qui résultent pour l'essentiel de la position de l'un des acteurs dominants, qui refuse de négocier de bonne foi avec l'ensemble des acteurs concernés. Je comprends donc parfaitement et partage le souhait de la commission de la culture du Sénat, inquiète de cette situation de blocage, de trouver une solution pour que ce droit voisin soit pleinement mis en oeuvre. La situation actuelle est néanmoins complexe et invite à la prudence. J'attire tout d'abord votre attention sur la nécessité d'agir avec précaution sur un plan juridique,

qu'une marge de manoeuvre très limitée. À cet égard, le Sénat s'est attaché à ce que la loi du 24 juillet 2019 soit aussi précise que possible, mais dans le strict respect du droit européen. En revanche, je ne suis pas convaincue que l'article 2 présente les mêmes garanties. Le vote d'une telle disposition pourrait susciter de nouveaux recours dilatoires de la part des plateformes et retarder encore la mise en oeuvre de ce droit voisin, auquel nous sommes très attachés. Par ailleurs, toutes les familles de presse, rejointes par l'Agence France Presse, ont déposé plainte contre Google- c'est de cette société qu'il s'agit ... -auprès de l'Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. La décision rendue par cette autorité le 9 avril 2020 conforte le bien-fondé de la demande des acteurs de la presse. L'Autorité de la concurrence devrait se prononcer très prochainement sur le respect par la société Google de l'injonction de négocier de bonne foi que l'Autorité lui avait adressée. Une nouvelle condamnation aurait nécessairement un effet décisif sur les négociations avec les éditeurs et les agences de presse. L'article 2 me paraît prématuré, dès lors que toutes ces voies de droit ne sont pas épuisées. tenu du contexte que je viens d'exposer, mon amendement vise donc à supprimer l'article 2 . Je veux cependant vous assurer, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, de l'engagement sans faille du Gouvernement à prendre toutes ses responsabilités dans les combats qu'il reste à mener sur ce sujet.

les négociations qui traînent en longueur ont contribué à fissurer le front des éditeurs et des agences, comme en a témoigné la table ronde édifiante organisée ici même par la commission le 14 avril Dans ce contexte, j'entends les réserves juridiques exprimées par Mme la ministre sur le dispositif de l'article 2 . J'observe cependant que d'autres pays, comme l'Australie, ont obtenu des résultats prometteurs sous la pression des pouvoirs publics. Dès lors, il me semble qu'il convient de bien marquer notre volonté de contraindre les grandes plateformes, non pas à recourir à des tactiques dilatoires, mais à négocier en toute bonne foi et avec la conscience aiguë qu'elles doivent respecter la volonté clairement exprimée des législateurs européens et nationaux. Nous attendons également, dans peu de temps, une décision de l'Autorité de la concurrence. La commission a entendu sa présidente, Mme de Silva, le 7 avril dernier : nous pensons qu'une prise de position ferme de sa part serait susceptible de faire bouger les lignes.

de la commission ? La lutte contre le piratage sportif est d'autant plus importante que les plateformes qui en profitent aujourd'hui ne sont pas situées en France et se rémunèrent en faisant payer les bénéficiaires.

J'ajoute à l'excellente démonstration du rapporteur un autre argument : la taxe adoptée sur l'initiative de Marie-George Buffet en 2000 garantit qu'une partie des droits de diffusion des manifestations sportives finance le sport amateur.

vise à mieux organiser un éventuel recours devant le juge en cas de difficulté d'application du mécanisme de notifications adressées par l'Arcom, sans pour autant laisser penser

Il me paraît absolument indispensable de confier à un magistrat l'exercice de la réponse graduée. Cela permet d'apporter toutes les garanties d'expertise et d'impartialité nécessaires à la mise en oeuvre de cette procédure de nature prépénale,

avec l'adoption future du. Cela justifie pleinement que le collège de l'Arcom puisse bénéficier de l'expertise de deux membres magistrats. Certes, la commission a souhaité entourer la mise en oeuvre de la réponse graduée de garanties particulières, en la confiant à un membre de l'Arcom « ayant une compétence juridique ». Cependant, la composition

des membres nommés par le Parlement, et la position de la commission, qui souhaite préserver l'influence du Parlement. Le compromis proposé prévoit de porter le nombre

À cette occasion, j'avais émis le souhait de conforter le rôle du service public dans la mise en valeur du sport à la télévision. J'avais envisagé plusieurs pistes pour atteindre cet objectif, notamment celle de distinguer, au sein du groupe France Télévisions, une chaîne référente en la matière. Les

ne remet pas en cause la stratégie globale et transversale de diffusion de contenus sportifs mise en place par France Télévisions et n'aurait pas pour effet de désinvestir France 2 et France 3 de la couverture des grands événements. En outre, cela serait complémentaire avec le développement de France TV Sport, désormais hébergé sur France Info.

Grâce à un travail itératif, sa rédaction a été améliorée afin de ne pas oublier Radio France, qui joue également un rôle important dans la diffusion de programmes sportifs. La place du sport sur le service public audiovisuel constitue un véritable enjeu, car son exposition est en baisse du fait de la hausse des droits de diffusion. Cet amendement a le mérite de poser la question de l'exposition du sport, même s'il ne règle pas la question des moyens. Le texte de la commission apporte déjà une réponse, puisque le maintien de France 4, seront destinés à la jeunesse en journée, ouvre la possibilité de consacrer les soirées alternativement à des programmes culturels et sportifs. Le présent amendement n'est aucunement contradictoire avec les objectifs de la commission : celle-ci partage le souci de réaffirmer la place du sport sur le service public. Par ailleurs, la notion de « services référents » présente l'avantage de n'empiéter ni sur le cahier des charges ni sur la liberté éditoriale des chaînes publiques, tout en réaffirmant un principe. Fallait-il prévoir cette disposition à l'article 43-11 ou à l'article 44

vous proposez de faire de l'une des chaînes de France Télévisions et de l'une des antennes de Radio France des « référentes » en matière de sport. n'y est pas favorable, d'abord pour une raison de principe tenant au périmètre du projet de loi : la redéfinition des missions de l'organisation du service public n'est pas l'objet du présent texte. Surtout, il ne me semble pas opportun de réserver l'exposition de programmes sportifs à une seule chaîne France Télévisions et Radio France jouent sur la complémentarité des chaînes qu'elles éditent pour offrir la meilleure exposition aux programmes qu'elles proposent. Elles déploient cette stratégie notamment en matière de diffusion du sport, qui est une composante essentielle de la mission de renforcement de la cohésion

C'est tout particulièrement le cas avec les vulgarisateurs et les vulgarisatrices historiques, qui éprouvent de grandes difficultés à traiter les sujets sensibles. On assiste donc à une forme d'autocensure par le revenu.

l'algorithme pratique assez largement la « surcensure ». Une nouvelle fois, les vulgarisateurs en sont les premières victimes et il est de plus en plus difficile de traiter de sujets comme la Seconde Guerre mondiale

de la commission ? Je partage l'objectif de cet amendement : protéger davantage les auteurs de contenus sur les plateformes. Pour autant, le dispositif proposé semble difficile à mettre en oeuvre, car il ne prévoit aucune sanction à l'encontre des plateformes qui ne joueraient pas le jeu du partage de la valeur.

et les droits voisins dans le marché unique numérique. Cette ordonnance comporte des dispositions qui permettront aux créateurs soit d'être rémunérés par les plateformes de partage qui diffusent leurs oeuvres, soit d'obtenir l'application de mesures préventives efficaces garantissant l'indisponibilité des contenus non autorisés. Ce faisant, l'ordonnance contribuera au partage de la valeur que vous appelez de vos voeux. elle apporte une plus grande sécurité juridique et de nouveaux droits au profit des utilisateurs. Les plateformes devront ainsi mettre en place un dispositif permettant aux utilisateurs de contester une situation de blocage ou de retrait d'une oeuvre mise en ligne ; si le litige persiste, ces derniers pourront introduire un recours devant l'Arcom.

il s'agit souvent de contenus cycliques qui participent à créer des dynamiques de vidéos, ainsi qu'une certaine uniformisation des contenus. Bien évidemment, les vidéastes ont leur responsabilité en la matière, car ce sont bien eux qui suivent la mode, mais on ne peut pas résumer la situation à ce seul exemple. Suivre les tendances, c'est être quasiment assuré d'être mis en avant, ce qui permet, outre la reconnaissance, d'engranger des vues et des interactions, donc des revenus. de revenus directs provenant de la plateforme en fonction du nombre de vues, mais aussi de revenus liés à des placements d'annonces avant, pendant et après les vidéos ou à des placements de produits au sein des vidéos, une certaine visibilité. Aussi, au vu de la place que prennent les algorithmes de mise en avant des plateformes, il semble normal qu'une certaine transparence soit appliquée. Nous aurions tort de laisser les plateformes s'autoréguler et surtout

littéralement l'internaute dans des contenus qui peuvent être de plus en plus négatifs. Il s'agit donc d'un sujet réel et important sur lequel j'espère que le futur régulateur aura à coeur de proposer une analyse globale. Quel est l'avis

La commission a souhaité garantir aux éditeurs un accès aux données relatives à la consommation de leurs programmes détenus par ceux qui les distribuent. Le Gouvernement partage l'objectif de favoriser l'accès des éditeurs à ces données, qui sont devenues indispensables à la connaissance des audiences et donc à la construction d'une grille de programmes correspondant aux attentes du public. Cependant, le principe d'un accès gratuit à ces données, dont la collecte suppose de la part des distributeurs des investissements conséquents, constitue à mes yeux une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Cela me paraît d'autant moins justifiable que la liberté contractuelle est aujourd'hui la règle s'agissant de la reprise des services par les distributeurs, qui fait parfois l'objet, d'ailleurs, d'une rémunération prévue dans le contrat. Je vous propose donc plutôt de confier la mission à l'Arcom de veiller à l'accès à ces données dans des conditions « équitables », sans imposer un principe de gratuité qui irait trop loin. En outre, je suggère

Concernant l'indépendance des médias, la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias avait précisément pour objectif de renforcer cette indépendance, la création des comités de déontologie en partant du principe qu'il n'était plus possible d'exercer un contrôle sur l'actionnariat. La commission, qui partage le constat fait par le gouvernement en 2016, émet un avis défavorable sur cet amendement.

le respect du principe de pluralisme des médias. Par cet amendement, il est proposé d'aller plus loin et d'interdire purement et simplement à des groupes opérant dans certains secteurs d'activité, au demeurant définis de manière très large, de détenir un service hertzien de télévision ou de radio.

des opérations de concentration n'aboutissent à une sorte d'hégémonie qui serait contraire au pluralisme et à l'indépendance.

est à M. Jérémy Bacchi. Il nous semble essentiel aujourd'hui de revoir notre copie. L'introduction dans la loi de 1986 dite Léotard d'un dispositif assurant la retransmission en clair de certains événements qualifiés d'importance majeure était une une bonne idée. Malheureusement, il a aujourd'hui atteint ses limites, non qu'il ne soit plus pertinent sur le fond, mais il se révèle insuffisant. À cet égard, les jeux Olympiques et Paralympiques sont révélateurs du problème. Lors des JO de Rio

Il faut d'ailleurs se rappeler que cette opération a été une bouffée d'air, car, entre l'obtention des droits par le géant états-unien en 2015 et l'accord conclu en 2019, a plané le risque que seules les 400 heures fixées par le CIO soient retransmises en clair. un autre exemple marquant, celui de la Ligue des champions de football. Il y a un peu moins de vingt ans, nous avons pu suivre sur TF1 l'épopée monégasque malheureusement achevée en finale contre Porto. Qu'en serait-il aujourd'hui ? Au vu de l'évolution du marché, alors que même la Coupe du monde n'est diffusée qu'à peine pour moitié en clair, on peut sérieusement craindre que ces événements de joie collective ne soient enlevés à tous les amateurs de sport.

au cyclisme, au handball et au tennis et un à la Formule 1 et à l'athlétisme, avec une forte prédominance pour le sport masculin. De la même manière, le handisport est totalement absent de la liste, les jeux Paralympiques n'étant même pas inscrits.

dont les droits télévisés ont été acquis par d'autres services. Néanmoins, on peut légitimement estimer que, entre la diffusion de ces brefs extraits et la diffusion exclusive des événements sur la base des droits attribués, il existe un créneau qui permettrait l'accès à un large public d'une information plus substantielle par la diffusion d'extraits un peu plus significatifs par des chaînes gratuites. À ce titre, cet amendement a pour objet la réservation à des chaînes gratuites par les ligues professionnelles, dans le cadre de la mise en vente de leurs droits audiovisuels, de lots consistant en un droit de diffusion d'extraits significatifs, et non brefs, de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires qui pourraient prendre la forme de magazines d'actualité. Ces supports permettraient d'assurer auprès du plus grand nombre la promotion de la pratique professionnelle de ces de ces disciplines en France. Dans de nombreux pays, les ligues professionnelles réservent ainsi à des chaînes gratuites un lot de magazines liés à leurs compétitions. C'est le cas de la première ligue anglaise, qui cède à la BBC les droits du magazine, institution de la institution de la télévision britannique diffusée depuis 1964. Cette proposition figurait dans le rapport que j'ai remis au gouvernement mais aussi dans le rapport d'information de l'Assemblée nationale du 3 juillet 2013 sur le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français.

commission ? L'amendement n° 49 rectifié vise à étendre de manière considérable les événements sportifs majeurs faisant l'objet d'une diffusion en clair, sans toutefois donner une liste précise ni évaluer le manque à gagner pour les fédérations, les ligues et les sociétés concernées. Si la situation actuelle n'est sans doute pas satisfaisante, il paraît judicieux de faire preuve de grande prudence en ce domaine, à un moment où le modèle économique des clubs, des ligues et des fédérations se trouve très fragilisé.

Si l'amendement n° 29 s'inscrit dans la même philosophie que les amendements n 27 rectifié et 28 rectifié, celle de permettre une meilleure visibilité du sport sur les chaînes en clair, il pose une difficulté supplémentaire, puisqu'il tend à créer une obligation pour les ligues professionnelles, alors que celles-ci rencontrent aujourd'hui des difficultés importantes pour vendre leurs droits. Une remise à plat du modèle économique des ligues professionnelles est sans doute nécessaire, mais il ne paraît pas opportun de créer aujourd'hui une contrainte supplémentaire, alors que, par exemple, la Ligue de football professionnel rencontre de sérieuses difficultés dans la vente de ses droits sportifs.

j'ai de nouveau contacté sur cette question, maintient que cet amendement est satisfait. Pour autant, dans la mesure où la rédaction proposée n'entre pas en conflit avec les prérogatives du régulateur, mais apporte peut-être une précision utile, je propose de demander l'avis du Gouvernement afin de mesurer l'impact exact de cette disposition.

remis un rapport d'une très grande qualité, à la suite d'une mission qui vous avait été confiée conjointement par la ministre de la culture, le ministre de la ville et le secrétaire d'État chargé des sports

dont les effets cumulés ont entraîné un véritable bouleversement du marché des droits audiovisuels sportifs, notamment ceux du football professionnel. Vous l'avouerez, ce contexte est peu propice

industries culturelles, avec l'ensemble des acteurs concernés des secteurs audiovisuel et sportif, en tenant compte de ce nouveau contexte. Pour l'instant, ces concertations se sont révélées

Par ailleurs, je peine à comprendre comment cette instance fonctionnerait : les diffuseurs sont en concurrence pour l'achat de droits sportifs et ne souhaitent pas nécessairement se coordonner, comme l'a montré l'achat des droits des jeux Olympiques de 2024 par France Télévisions au prix fort, alors que TF1 et M6 étaient prêtes à partager le fardeau. Le CSA ne pourra donc pas coordonner des stratégies d'entreprise qui divergent, ce n'est pas son rôle. La

et ce de manière homogène sur tous les téléviseurs, indépendamment des modalités de diffusion ou de réception. Ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui en France, où la compatibilité des téléviseurs avec ces services interactifs est très imparfaite. À l'inverse, on constate que les téléviseurs sont systématiquement compatibles avec les grandes plateformes américaines de vidéo à la demande ; celles-ci y sont préinstallées dans le cadre d'accords mondiaux avec les constructeurs, ce qui leur donne un avantage considérable de visibilité et de diffusion. Il faut remédier, par une obligation de compatibilité des téléviseurs, à cette situation qui pénalise les Français et les éditeurs nationaux et compromet lourdement notre souveraineté culturelle.

au bouquet des programmes de la TNT : guide des programmes de la TNT, portail permettant d'accéder à des contenus à la demande, etc. Cela est indispensable pour maintenir l'homogénéité et la continuité de l'offre entre la TNT et les autres réseaux.

rectifié vise à étendre aux services interactifs émis par un éditeur de la TNT le principe de l'intégrité du signal récemment ajouté à la loi par l'ordonnance de transposition de la directive SMA. Il est satisfait par le 1° de l'amendement n° 96 que j'ai déposé et qui pose le principe de la nécessité d'un accord des éditeurs pour modifier la signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle. Le sujet est extrêmement important ; il s'agit de renforcer l'attractivité de la plateforme TNT.

D'une part, de telles obligations de compatibilité des téléviseurs à l'interactivité sont difficilement conciliables avec le droit communautaire en matière de libre circulation des marchandises. Ce cadre ne permet d'imposer aux téléviseurs que des exigences dites Il s'agit par exemple d'obligations permettant une utilisation plus efficace des ressources en fréquence, ce qui est notamment le cas des obligations de compatibilité proposées à l'amendement n° 1 Une obligation de compatibilité des téléviseurs à la technologie Hbb TV est d'autant plus discutable que les fabricants lui dénient à ce jour son statut de norme européenne.

Je suis sensible à votre demande, mais attendons que le bilan des expérimentations en cours ait confirmé les espoirs que nous plaçons en cette technologie. Je m'engage à conforter la place du Hbb TV dans l'écosystème de la TNT, en préparant une modification de l'arrêté dit signal en lien étroit avec les éditeurs et les fabricants.

et à venir dans le cadre du bouquet de chaînes correspondant à son mode de réception. Le guide de programmes de la TNT doit ainsi rester dans l'environnement TNT, au risque d'apporter une information erronée aux téléspectateurs ou de faire doublon avec les guides électroniques de programmes proposés par les distributeurs.

Le scandale Mediapro n'est que la conclusion inéluctable d'années, voire de décennies, d'errance : une minorité d'acteurs a tenté de se tailler une grosse part du gâteau, quitte à faire prendre des risques à tous les autres.

se positionner sur la bulle des droits télévisés, des transferts et des salaires, le sport étant un marché concurrentiel. Aujourd'hui, son soutien serait nécessaire. La dérégulation engagée depuis des décennies n'aurait-elle donc pas que

la grande majorité des pirates sont justement des supporters qui n'ont plus forcément les moyens financiers, pratiques, voire légaux, d'aller au stade ou de prendre des abonnements télévisés pour suivre leur équipe. Finalement, c'est tout l'écosystème du sport professionnel mis en place au cours de ces dernières années qui devra être revu pour lutter contre le piratage.

activement accompagné la naissance et le lancement en 2005. Quinze ans plus tard, l'heure est venue de franchir une nouvelle étape, en lançant les services TNT en ultra haute définition (UHD) pour une meilleure qualité et un meilleur rendu. Cela implique évidemment de nouvelles obligations en matière de compatibilité des récepteurs de télévision. Je ne saurais trop insister sur les nombreux atouts de la TNT. D'abord, la couverture est large : plus de 97 % de la population à l'échelle nationale,

sur deux. Il est important de légiférer pour apporter de nouveaux outils au régulateur afin de réaliser une transition qui conciliera l'intérêt de l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel l'audiovisuel et de répondre aux attentes des téléspectateurs en matière d'amélioration de la qualité de la diffusion hertzienne terrestre. Il s'agit évidemment d'une expérimentation. Elle devra être évaluée et suivie de près par le CSA, qui a déjà réfléchi à un programme de travail précis et à des étapes successives à franchir. Il me semble important de ne pas laisser passer le train de la modernité, surtout au regard des défis que nous devrons relever. Ainsi, dans la perspective des jeux Olympiques de 2024,

la phase d'expérimentation, qui devrait s'achever en 2024 ou 2025. L'ensemble des chaînes de la TNT pourront-elles alors basculer en UHD ? Faudra-t-il se résoudre à faire coexister des chaînes en haute définition et d'autres en ultra haute définition ? Quel sera le coût de cette technologie pour les foyers français, pour les chaînes et pour les producteurs de programmes ? Existe-t-il un risque que certaines « petites » chaînes se retrouvent exclues de la plateforme TNT pour permettre aux grandes chaînes d'émettre à

dont l'examen a été interrompu au mois de mars 2020. Pour des raisons tenant aux contraintes du calendrier parlementaire, j'ai fait le choix, difficile, de renoncer à ce volet dans le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui. Mais je partage votre attachement constant à la TNT, qui demeure le seul moyen d'accès à la télévision de plus d'un foyer sur cinq dans notre pays et qui reste utilisée par un foyer sur deux. Si vos propositions me paraissent excéder le périmètre du présent projet de loi,

publique, a établi un programme et fixé des perspectives. Il est bien naturel de lui demander d'évaluer l'expérimentation pour pouvoir se projeter utilement.

peu diffusés, moins connus, qui ont pourtant, parfois, beaucoup d'adeptes et de pratiquants. Et je pense évidemment aussi au sport féminin.

a introduit la possibilité pour l'Arcom de reconduire une seconde fois, hors appel à candidatures, les autorisations délivrées aux chaînes de la TNT, pour une période de cinq ans. Le fort risque

d'abord que le régime de la double reconduction a déjà existé pour les chaînes de télévision entre 1986 et 2002 et existe toujours pour les services de radio. Il est donc bien conforme aux règles de protection du domaine public. Le motif d'intérêt général qui légitime la réintroduction d'un second renouvellement est par ailleurs constitué par la nécessité de préserver l'attractivité de la plateforme TNT, sur laquelle pèsent, qu'on le veuille ou non, des

Le Gouvernement est favorable aux modifications apportées par la commission au régime obligeant les distributeurs de services à reprendre les chaînes de service public. Je souhaite toutefois y apporter deux précisions. d'une part, d'étendre ces garanties nouvelles aux chaînes publiques locales. Ces services d'initiative publique locale consacrés aux informations sur la vie locale bénéficient aussi de cette obligation de reprise, et il m'apparaît donc normal de leur appliquer la garantie de conclusion d'un contrat que vous avez introduite. Je propose, d'autre part, de supprimer la garantie de reprise des programmes de service public de manière simultanée, en intégralité et sans altération, cette garantie étant déjà assurée pour tous les services

est à M. le rapporteur. Il résulte de l'observation de la pratique des distributeurs que, lorsque ces derniers reprennent au sein de leur offre de services des chaînes de la TNT à vocation locale

en haute définition, d'autres non. Une telle dégradation du signal est également susceptible de porter atteinte à la visibilité des chaînes de la TNT à vocation locale et au confort d'utilisation du téléspectateur.

le périmètre du texte et il pourrait soulever des difficultés pratiques. Il ne faudrait pas qu'il ait pour effet paradoxal d'empêcher les fournisseurs d'accès de proposer, en accord avec les éditeurs, des formats de diffusion encore meilleurs que la HD-

prévu par la loi Léotard pour éviter les phénomènes de concentration. Alors que le secteur des médias et de l'audiovisuel a déjà fait l'objet d'opérations de rachat et de concentration, il n'apparaît pas opportun d'élargir encore de telles possibilités. Au moment où les discours médiatiques sont de plus en plus plus en plus remis en cause et où la lutte contre les fausses informations doit être une priorité, il est contradictoire de favoriser le rassemblement de groupes audiovisuels et l'uniformisation des lignes éditoriales. Si l'arrivée des plateformes numériques inquiète légitimement, il est vain de penser que le simple regroupement des entreprises audiovisuelles leur donnera la puissance économique de venir rivaliser avec elles. Cela ne pourra qu'entraîner une nouvelle vague d'uniformisation des programmes et des lignes et des lignes éditoriales. Enfin, l'existence de dispositifs poussés de coopération comme Salto démontre la capacité des acteurs de l'audiovisuel de s'allier. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. La parole est à M. Jean-Pierre

Le relèvement du plafond de couverture applicable aux télévisions locales de 12 à 30 millions d'habitants, comme le prévoit l'amendement adopté en commission, devenu

pourrait ouvrir la voie à une concentration excessive dans le secteur. Un relèvement du seuil à 30 millions permettrait en effet au même groupe de couvrir, par les chaînes locales qu'il détient, une population avoisinant les deux tiers de la population française.

30 septembre 1986, afin de porter de 12 millions à 30 millions d'habitants le seuil anti-concentration pour les réseaux de télévision locale. Il porte le risque d'une déstabilisation du secteur.

et le travail menés depuis une semaine- rien ne sort du chapeau, monsieur Assouline -ont permis de considérer que le seuil de 20 millions d'habitants était sans doute plus adapté pour concilier le développement nécessaire de certains réseaux et la nécessité de préserver les chaînes locales existantes. C'est la raison pour laquelle je donne un avis favorable sur l'amendement

n'est pas de reconstituer un réseau national. Pour cela, il est proposé d'ajouter un critère de différenciation à hauteur de 80 % des programmes originaux et locaux sur chaque chaîne du réseau détenu par un même groupe.

être satisfaite par un réseau de chaînes d'information, elle pourrait en revanche ne pas être tenable pour un réseau de chaînes généralistes ou culturelles. On peut comprendre l'objectif de cet amendement, qui est de renforcer la dimension locale des chaînes faisant partie

Cet amendement tend à donner la possibilité légale aux organismes de gestion collective de saisir l'Arcom du non-respect, par les éditeurs et distributeurs de services,

Cette décision précise que, « indépendamment des organisations et associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, s'agissant des sociétés du secteur public de la radio et de la télévision, et au dernier alinéa de l'article 42 de la même loi, s'agissant des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des opérateurs de réseaux satellitaires, toute personne qui dénonce un comportement d'un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure ». Néanmoins, l'ajout dans la loi des organismes de gestion collective reste une nécessité, pour au moins deux raisons.

de la commission ? Nous avons débattu de cet amendement en commission et j'avais proposé à son auteur de le déposer en séance, ce qu'il fait aujourd'hui, afin d'obtenir des garanties de Mme la ministre.

1997. D'autre part, une autre décision, plus récente, du Conseil d'État- elle date du 7 février 2017 -a relativisé la portée de la liste établie à l'article 42 dorénavant, toute personne dénonçant un comportement d'un opérateur qui porte atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure. En conséquence, il semble assuré que les organismes de gestion collective ont dorénavant toute faculté pour saisir le CSA et, demain, l'Arcom.

les organismes mentionnés à l'article 42 de la loi de 1986 incluent bien ces organisations. J'observe d'ailleurs que la SACD a déjà mis en oeuvre cette faculté, comme l'a rappelé M. le rapporteur. La jurisprudence du Conseil d'État est encore plus large,

nécessaire d'être inscrit sur la liste de l'article 42 pour pouvoir demander au CSA de prononcer une mise en demeure ; il suffit de justifier d'un intérêt à agir et tel est, naturellement, le cas des organismes de gestion collective. Nous n'avons donc pas de désaccord sur le fond,

de la loi de 1986 pour prévoir l'association des auteurs aux négociations professionnelles, en jugeant utile de préciser qu'il s'agit « des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs

les accords doivent être conclus « entre les organismes professionnels d'auteurs, les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie [et] les organisations professionnelles représentatives des producteurs ». Cet amendement

Cet amendement tend à permettre à l'autorité de régulation d'appliquer, sans que sa décision et le fondement de celle-ci puissent être contestés, le retrait ou la résiliation de l'autorisation d'un service, lorsque l'opérateur aura diffusé un programme contenant des propos d'incitation à la haine.

qui n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire définitive. J'ajoute que le CSA ne demande pas de disposer d'un tel pouvoir ; je remarque en outre que le renouvellement des autorisations peut également permettre de renforcer, au besoin, les engagements des chaînes dans la lutte contre les propos haineux. La commission a donc émis un avis

Je parle d'une émission dont l'éditeur connaît le contenu avant sa diffusion, puisqu'elle est enregistrée une demi-heure avant. Dans cette émission, ce n'est pas un invité qui dérape, c'est quelqu'un qui est payé pour déraper

et que, si l'on n'y fait pas attention, si l'on considère que ce n'est rien, il va bientôt nous tomber sur la tête de graves désagréments. J'aurai au moins posé le débat et je prends date.

présent amendement vise à rééquilibrer l'article 13, qui relève le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d'être infligées par la future autorité de régulation et applicables dans le cas spécifique des manquements relatifs aux obligations de financement, par les éditeurs, de la production audiovisuelle et cinématographique.

mais sur leur assiette totale -et, d'autre part, des niveaux de sanction maximale auxquels peuvent recourir les autres autorités administratives indépendantes comparables au CSA, fondés sur un pourcentage de chiffre d'affaires. Il en ressort un caractère manifestement disproportionné des sanctions au regard de la nature du manquement, ce qui rend cette disposition potentiellement confiscatoire pour des éditeurs nationaux dont la situation financière est sans commune mesure avec celle d'acteurs mondialisés, certes soumis au même cadre depuis l'ordonnance du 21 décembre 2020, mais pour lesquels l'impact économique de ce nouveau régime de sanction serait infiniment moindre. Afin de préserver la logique d'équité et de proportionnalité revendiquée dans le projet de loi, il est proposé d'aménager la rédaction de ce nouveau régime, en renvoyant explicitement la sanction pécuniaire qui lui est rattachée, ainsi que le relèvement du plafond y afférent, au manquement constaté par rapport aux obligations visées,

potentiellement très significatif de l'amende pouvant être infligée à l'éditeur. Il met en avant la différence de l'impact d'une telle sanction pour un éditeur national et pour les grandes plateformes mondialisées, qui pourraient beaucoup plus facilement l'absorber.

le Conseil d'État a ainsi admis un quadruplement du barème du tarif publicitaire. La disposition prévue par cet amendement constituerait un recul par rapport à cette jurisprudence, en limitant le plafond de la sanction au double du montant du manquement. je ne partage pas votre jugement sur le caractère disproportionné de la sanction proposée à l'article 13 du projet de loi. Je le rappelle, cette sanction, fixée au double du montant de l'obligation, est un plafond que le CSA ne peut dépasser ; il peut donc évidemment fixer un montant moins élevé. le CSA adaptera la sanction pécuniaire à la gravité du manquement, sous le contrôle du juge. Si les investissements de l'éditeur dans la production sont légèrement inférieurs à son obligation de contribution, la sanction sera évidemment plus faible que si l'éditeur a totalement méconnu

pour les services en ligne. D'ores et déjà, un certain nombre de conventions conclues entre les opérateurs de l'audiovisuel et le CSA prévoient expressément le respect des droits d'auteur. De la même manière, l'autorité de régulation a eu l'occasion d'intervenir dans des conflits récents autour des manquements de certains éditeurs à l'égard des droits d'auteur.

si l'on y regarde de plus près, le désamour d'une partie du public pour la télévision tient au sentiment d'un manque d'audace des programmes. Ce n'est donc pas en uniformisant un peu plus encore les contenus et les discours qu'on luttera contre ce phénomène. Il ne nous paraît donc pas opportun de faciliter ce genre d'opération.

l'article 13 , introduit par votre commission. À plusieurs reprises, au cours des dernières années, le législateur et le Gouvernement ont pris des mesures pour lutter contre les pratiques spéculatives en matière d'attribution et de cession d'autorisations d'occupation du domaine public hertzien. Les fréquences sont un bien rare du domaine public de l'État ; elles sont attribuées, depuis 1986, après une procédure d'appel à candidatures. Nous avons tous été choqués de la pratique de certains opérateurs, qui ont revendu leur société peu de temps après avoir été autorisés à émettre, alors qu'ils nous avaient promis monts et merveilles en matière de programmation pour obtenir depuis une modification apportée en 2016, l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 prohibe le changement de contrôle des services de télévision de la TNT pendant un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, sauf en cas de difficultés économiques qui menaceraient la viabilité de la société. Votre commission a proposé de déroger à ce principe pour les services qui ont bénéficié d'une première autorisation et qui en obtiendraient une nouvelle. Le Gouvernement n'est pas favorable à une telle dérogation ; une chaîne qui postule à l'obtention d'une autorisation, qu'il s'agisse d'une première autorisation ou d'un renouvellement, doit s'engager à exploiter la fréquence à laquelle elle prétend pendant une durée minimale. Quel est l'avis de la

dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques. Cette disposition visait à lutter contre la spéculation sur les reventes de fréquences- Mme la ministre vient de 2016, fait au nom de la commission de la culture, notre collègue Catherine Morin-Desailly s'interrogeait déjà « sur la nécessité d'adopter une disposition générale qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer les décisions économiques qui ne relèvent pas de démarches spéculatives ». Ce risque semble aujourd'hui réel, dans un contexte marqué par une restructuration du secteur des médias provoquée par la montée en puissance irrésistible des plateformes numériques américaines. Dans ces conditions, l'article adopté par la commission corrige la rédaction de l'article 42-3 de la loi de 1986, en excluant explicitement du dispositif les sociétés qui auraient déjà exploité des autorisations d'émettre, en application de l'article 30-1

Le dispositif de l'avant-projet de loi a été modifié de manière substantielle, après l'examen du texte par le Conseil d'État, lequel avait estimé que le dispositif initialement prévu d'autorisation préalable du ministère, lors de la cession d'un catalogue français, pouvait porter atteinte au droit de propriété et au principe de libre circulation des capitaux issu du droit européen et que les atteintes susceptibles d'être portées à l'intégrité, à la diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel,

notamment de la part d'acquéreurs étrangers qui peuvent très bien avoir intérêt à acheter un catalogue pour valoriser un titre et à laisser ensuite en déshérence, dans l'oubli et sans entretien, le reste du catalogue.

est à Mme Laure Darcos. Aux termes du dispositif prévu par l'article 17 du projet de loi, c'est bien au producteur cédant qu'incombe l'obligation de notifier au ministre chargé de la culture la cession de l'oeuvre ou l'opération équivalant à une cession. C'est également le producteur cédant que le ministre chargé de la culture informe de la saisine de la commission de protection de l'accès aux oeuvres. Enfin, c'est à son encontre que le même ministre peut prononcer une sanction pécuniaire en cas de manquement à l'obligation de notification de la cession. Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que le cédant et non le cessionnaire est visé dans ces trois étapes du dispositif.

il importe que les délais de réalisation de l'opération ne soient pas allongés de manière excessive et demeurent conformes aux pratiques du monde des affaires. Le présent amendement propose de ramener à trois mois au lieu de six le délai s'écoulant entre la notification au ministre chargé de la culture et la date prévue pour la réalisation de l'opération. Il réduit également à deux mois le délai durant lequel le ministre se prononce sur l'opération.

cette terminologie est donc loin d'être anodine. Il semble préférable de désigner explicitement « l'acquéreur des oeuvres », terme bien plus précis qui permet de lever toute confusion. L'amendement n° 47,

au titre du dépôt légal. Cela nous aurait permis de bénéficier d'un catalogue public de plus en plus riche, sans léser les producteurs. Malheureusement, comme le mentionne l'étude d'impact du projet de loi, les moyens d'action du CNC demeurent limités. Doter l'établissement de prérogatives de nature à lui permettre de procéder à l'acquisition de catalogues très importants, soit en volume, soit en valeur, serait disproportionné sur le plan budgétaire et technique en raison des moyens requis pour une telle entreprise. On aurait aussi pu instaurer un régime de déclaration préalable et d'autorisation, comme nos collègues socialistes l'ont proposé. Cela aurait été une protection supplémentaire des catalogues, mais aussi des spectateurs. Une nouvelle fois, cette idée, qui était celle du Gouvernement dans la première mouture du texte, a été repoussée par le Conseil d'État qui a considéré cette atteinte aux libertés contractuelle disproportionnée.

: La parole est à Mme la ministre. L'amendement n° 79 précise que le délai d'instruction d'un dossier par la commission de protection de l'accès aux oeuvres constitue un délai maximum et non impératif. Il va de soi que, lorsque les dossiers ne posent pas de problème, la commission n'a pas à être saisie.

à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. Le présent sous-amendement réduit ce délai à un mois, ce qui me semble suffisant pour permettre à la commission d'organiser la procédure d'instruction contradictoire, d'entendre les parties à l'opération et de rendre son avis.

se lire en complément de l'amendement n° 22. J'ai peur, hélas, que les mesures très contraignantes proposées dans cet amendement ne se heurtent aux remarques du Conseil d'État sur l'avant-projet de loi et au respect des droits de propriété des producteurs. Il s'agit, dans le cas d'espèce, d'une réelle limitation de leurs droits patrimoniaux, qui ne me paraît pas conforme aux règles de droit. La commission a donc émis un avis défavorable de l'amendement n° 22, le régime d'autorisation préalable envisagé pour les résidents de l'espace économique européen semble identique à celui des non-résidents.

l'amendement n° 9 rectifié, il paraît légitime de ne pas trop contrarier la vie des affaires avec des délais trop longs. Néanmoins, il faut aussi que la décision du ministre de la culture soit prise de manière éclairée. Aussi, je propose d'entendre l'avis du Gouvernement pour savoir si les conditions proposées par Laure Darcos sont réalistes pour les services du ministère. L'amendement n° 23 rectifié

l'amendement n° 47, la formulation retenue par ses auteurs traduit le souci que les oeuvres demeurent accessibles à des conditions tarifaires raisonnables. Nous ne pouvons que partager cet objectif s'agissant d'oeuvres patrimoniales. La rédaction retenue est relativement peu contraignante- il serait, au demeurant, difficile d'aller au-delà, s'agissant de droits de propriété. Je souhaite, toutefois, en savoir plus sur les conséquences concrètes de cette proposition sur l'examen auquel devra se livrer le ministère. Dès lors, je sollicite l'avis du Gouvernement.

: un régime déclaratif, lorsque le cessionnaire exerce son activité à l'intérieur de l'espace économique européen, et un régime d'autorisation, lorsqu'il exerce son activité en dehors de cet espace. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de liberté de circulation des capitaux,

à remplacer, par un dispositif d'autorisation préalable, celui de simple notification préalable des transferts de propriété d'un catalogue aux personnes non soumises à l'obligation d'exploitation suivie. suivie. Le Conseil d'État a estimé qu'un dispositif d'autorisation, comme le Gouvernement l'avait initialement envisagé, était notamment incompatible avec l'interdiction du contrôle des investissements étrangers, formellement prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cet amendement permet de lever toute ambiguïté sur l'application du dispositif. L'amendement n° 9 rectifié vise à réduire les délais de notification préalable et de la procédure devant le ministre chargé de la culture, chargé de la culture, réduisant à trois mois le délai de notification préalable de l'opération et à un mois le délai dont dispose le ministre de la culture pour se prononcer. L'amendement n° 72 que j'ai présenté clarifie déjà le délai d'instruction d'un dossier par le ministère de la culture, en précisant que la décision est rendue « sans délai », lorsque les garanties de recherche d'exploitation suivie sont suffisantes. Les trois mois que l'amendement tend à imposer peuvent être insuffisants

est défavorable à cet amendement qui crée une ambiguïté sur les opérations soumises au mécanisme de notification préalable. Je rappelle que l'article 17 vise les cessions et toutes les opérations d'effet d'effet équivalent. La notion de « bénéficiaire de l'opération » est donc plus large que la notion d'« acquéreurs des oeuvres » qui s'applique aux seules cessions. Il faut la conserver pour prévenir les risques de contournement de la procédure par des montages financiers sophistiqués. Monsieur Assouline,

est évident que l'accès du public aux oeuvres est un objectif de politique publique essentiel ; toutefois, les conditions tarifaires dans lesquelles seront exploitées les oeuvres cédées ne sont pas du tout déterminées lors de la cession de l'oeuvre, qui ne porte pas sur son exploitation, mais sur sa propriété. L'obligation de recherche d'exploitation suivie ne prévoit, par ailleurs, aucun critère tarifaire. Il ne peut donc pas y avoir un critère tarifaire dans la notification au ministre de la cession par un producteur d'une ou plusieurs oeuvres ou de toute autre opération assimilée.

Gouvernement clarifie le délai d'instruction d'un dossier par la commission de protection de l'accès aux oeuvres et permet déjà, en précisant que les trois mois de procédure sont un maximum, que la commission statue plus vite dans les cas les plus faciles. Pour cette raison, le

de la commission ? On ne peut que partager l'objectif de cet amendement qui vise à rappeler que les programmes dédiés à la jeunesse sur la chaîne publique qui lui est consacrée doivent respecter les objectifs de qualité, de diversité et d'équilibre entre contenus éducatifs et contenus divertissants. Toutefois, il paraît difficile d'ajouter ces précisions dans un alinéa qui est d'abord consacré au cahier des charges de France Télévisions, sauf à en changer l'équilibre. Par Par ailleurs, l'amendement tend à insérer une nouvelle phrase pour évoquer l'absence de publicité au lieu de garder cette précision dans la même phrase, ce qui pourrait avoir pour effet de signifier que l'ensemble des chaînes visées par le cahier des charges de France Télévisions est dépourvu de publicité. Le rapporteur serait favorable à cette évolution, mais il est évident qu'elle dépasse l'objet de ce texte et sans doute même l'intention de l'auteur. La commission a donc émis un avis

La réforme du régime de contribution à la production est, en effet, entamée depuis plusieurs mois. Elle doit se traduire par une modification des dispositions applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), ainsi qu'aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (TNT) et sur les autres

et de rééquilibrer les obligations des acteurs historiques et des nouveaux entrants selon une logique d'équité. Cette réforme globale est en voie de finalisation. Le projet de décret relatif aux SMAD a fait l'objet d'un avis du CSA et a été examiné par le Conseil d'État. le décret TNT, les diffuseurs et les organisations professionnelles de l'audiovisuel et du cinéma ont négocié pendant quatre mois, jusqu'à fin avril, et le Gouvernement s'apprête à présenter sur cette base un projet de décret révisé. Compte tenu de la cohérence d'ensemble qui unit ces différents volets, le Gouvernement souhaite que ces décrets soient stabilisés de manière simultanée, d'ici à la fin du mois de juin. Une modification du cadre législatif, en particulier de la définition de la production indépendante en matière audiovisuelle, risque de bouleverser ce calendrier, de perturber les discussions en cours et, finalement, de retarder l'entrée en vigueur de la réforme, très attendue par l'ensemble des professionnels. En outre, la simplification proposée pourrait avoir pour effet d'interdire au pouvoir réglementaire d'encadrer, au sein de la part indépendante des chaînes hertziennes, les parts de coproduction et les mandats. Cela créerait une asymétrie entre le décret TNT et le décret SMAD,

pire, de remettre en cause l'aboutissement imminent des discussions sur le décret TNT. Bacchi, pour présenter l'amendement n° 89. L'éventail des relations entre les producteurs et les éditeurs de services va globalement de la courtoisie, au mieux, à la conflictualité dure, au pire. Dans ce cadre, et alors que les producteurs et les éditeurs audiovisuels sont en pleine concertation avec le ministère pour

de la commission ? Le Gouvernement justifie la demande de suppression de l'article 17 par la nécessité de conduire à son terme la négociation sur le décret TNT. À notre connaissance, cette négociation est aujourd'hui dans l'impasse ! Le projet de décret présenté cette semaine aux parties concernées comprend une baisse très faible du taux d'indépendance, qui ne change pas la situation des chaînes gratuites, ainsi qu'une refonte du régime de Canal+ qui pourrait porter préjudice à ce groupe. L'accès aux parts de coproduction serait également assoupli à la marge, lorsque le producteur finance la moitié du devis, ce qui ne répond que partiellement au problème de France Télévisions, par exemple. Face à ces ajustements mineurs, il nous revient que les autres critères de l'indépendance seraient renforcés, comme la durée des droits, ce qui ne saurait répondre aux besoins des diffuseurs qui doivent pouvoir exposer durablement leurs contenus sur plusieurs supports. Le rapport Le rapport de notre collègue Jean-Pierre Plancade avait mis en évidence, dès 2013, le fait que les règles qui définissent le régime de la production, fixées en 1986, n'étaient plus adaptées, ce que l'on peut Or, avec l'arrivée des plateformes, la position défavorable des chaînes n'a fait que s'accentuer dangereusement. Concernant en particulier le service public de l'audiovisuel, il est devenu incompréhensible que France Télévisions, qui dépense près de 500 millions d'euros dans la création, ne puisse pas valoriser cet investissement ni sous la forme de mandats, lorsque les producteurs sont dépourvus de capacité de distribution, ni à travers des parts de coproduction sur l'animation et le documentaire, comme l'indiquent les données transmises par l'entreprise et publiées dans le rapport À maints égards, comme je l'ai déjà indiqué, la contribution à l'audiovisuel public est devenue une contribution à la production privée ! Le législateur est dans son rôle, en faisant évoluer un principe ; il conviendra aux parties prenantes de s'adapter en conséquence.

à laquelle elle se rattache, en disposant que « chaque assemblée [dote] sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions ». Afin de permettre à ces chaînes de disposer de ressources complémentaires, le présent amendement vise à les autoriser à percevoir, à titre accessoire, des revenus provenant de l'exploitation des programmes audiovisuels dont elles assurent la production et la réalisation. Cette rédaction permet de préserver le principe d'un financement

Il est important que la totalité de nos concitoyens y ait accès dans des conditions respectueuses du droit d'auteur et des droits voisins. C'est pourquoi la loi de 1986, telle que modifiée par la loi du 14 octobre 2015, dispose que « les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain » et que, « à cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements. Néanmoins, force est de reconnaître que le code de la propriété intellectuelle n'a pas été modifié de façon à tirer explicitement les conséquences de modes particuliers de diffusion des chaînes de la TNT en clair. Conformément à l'article 98-1 de la loi de 1986, il existe des offres de diffusion par satellite des chaînes de la TNT en clair, qui ne demandent aux téléspectateurs aucun abonnement. Elles ne touchent pas non plus de rémunération de la part des chaînes. Le modèle économique de ces offres, défini par la loi, ne permet pas à leurs prestataires de supporter des coûts au titre du droit d'auteur et des droits voisins. Ces services offrent aux chaînes hertziennes en clair un complément significatif de couverture : jusqu'à 20 % de la population dans certains départements, pour un total de l'ordre de 4 millions de foyers en France métropolitaine. C'est par exemple le cas de la Corse, avec 20 %, ou de la Vendée, avec 16 %. Cette diffusion satellitaire permet aux chaînes TNT, détentrices en amont des autorisations des sociétés d'auteurs, d'exécuter leur obligation de diffusion sur l'intégralité du territoire français.

Pour toutes ces raisons, il convient de considérer que les opérateurs des offres satellitaires répondant aux conditions de l'article 98-1 de la loi de 1986 ne réalisent pas une représentation supplémentaire et ne sont pas redevables de rémunérations au titre du code de la propriété intellectuelle. Faute d'une telle clarification, les offres de TNT gratuite par satellite pourraient disparaître, au détriment de nos concitoyens, en particulier les plus modestes, situés en zone blanche ou grise de la diffusion hertzienne terrestre. de la commission ? Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la diffusion de chaînes de la TNT sans abonnement par satellite. Cette diffusion ne créant pas de revenus pour le diffuseur satellitaire, il est difficile de considérer qu'elle puisse créer une charge au titre du droit d'auteur et des droits voisins.

de radio, dite CabSat 2, que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne prévoient que, lorsque les distributeurs de signaux se limitent à fournir des moyens techniques aux éditeurs, ils ne sont pas considérés comme participant à un acte de communication au public. Les opérateurs satellitaires répondent à cette condition, puisqu'ils fournissent uniquement un moyen technique permettant de garantir la réception de signaux. Si les opérateurs satellitaires n'ont donc pas de raison d'être mis à contribution dans ce cadre, cela ne signifie pas pour autant que les éditeurs ne doivent pas être interrogés concernant cette forme de diffusion de leurs programmes. Peut-être convient-il d'apporter des précisions quant au paiement des redevances réclamées aux opérateurs satellitaires.

Je ne suis pas d'accord avec votre analyse juridique, monsieur le rapporteur : cette disposition constituerait une exception au droit d'auteur et n'est donc pas conforme aux textes européens applicables en la matière. Pour autant, il me paraît essentiel que la diffusion des programmes des chaînes gratuites de la TNT puisse être assurée dans les zones dites blanches. Je vous annonce donc le lancement, dans les prochains jours, d'une mission de médiation entre les diffuseurs et les ayants droit concernés. Cette médiation devra s'efforcer de trouver une solution qui garantisse la rémunération légitime des auteurs, tout en tenant compte de l'objectif de couverture du territoire national. Je sollicite donc

Céline Boulay-Espéronnier, mais je suis entièrement d'accord avec Mme la ministre. Je suis bien évidemment favorable aux activités des opérateurs satellitaires qui procèdent à la retransmission de tous les programmes

qui utilise un mode technique spécifique doit être autorisée par l'auteur de cette oeuvre. Par conséquent, une mise à disposition des oeuvres par le biais de la retransmission par satellite d'une radiodiffusion télévisuelle terrestre

Les articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 avaient trait à l'acquisition des actions de la société nationale de programme TF1 lors de sa privatisation. L'article 22 de l'ordonnance du 21 décembre 2020,

de loi tend à supprimer leur mention. Toutefois, l'imposition prévue par cet article est toujours susceptible de s'appliquer lors d'une éventuelle cession de titres de la société TF1. Il convient donc de corriger le texte afin de maintenir

structure qui les emploie, ce qui pose des questions pour la reconnaissance de leurs droits. Parmi ces droits figure la rémunération proportionnelle aux résultats. En l'état, comment justifier de la participation d'un artiste au projet ? De la même manière, au vu de la multiplication des formes de contrats très courts dans le secteur culturel, cette inscription fait office de justificatif de travail. Il est donc proposé que l'ensemble des artistes soit mentionné au générique afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Quel est l'avis de la commission ? Il s'agit

Ce droit est déjà reconnu par le code de la propriété intellectuelle, y compris dans le secteur des oeuvres audiovisuelles. Au reste, la rédaction de l'amendement me pose problème, parce qu'elle n'impose la mention du nom des auteurs que sur les supports d'exploitation des oeuvres. Or cette mention du nom s'impose également, lorsque les oeuvres sont exploitées de manière dématérialisée,

public audiovisuel. Cet objectif fait d'ailleurs sens, alors que le Gouvernement a fait de la lutte contre les fausses informations une priorité. Il se trouve que le canal 19 va certainement se libérer.

pour une durée de trois mois seulement, ne me paraît pas opportun. En effet, la durée de trois mois ne sera pas suffisante pour permettre, d'une part, au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires qu'impose la mise en oeuvre de cette mission, et, d'autre part, à la Hadopi de mobiliser l'ensemble des moyens humains et matériels requis. Je vous propose donc la suppression de cet article, tout en vous confirmant l'engagement du Gouvernement en faveur d'une mise en place rapide de l'Arcom.

à la télévision d'information du service public d'être un peu plus proche des chaînes concurrentes.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, deux jours après mon arrivée en responsabilité au ministère de la culture, j'étais devant vous pour solliciter votre

modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique. Nous passons

de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.